La procédure accélérée a été engagée sur ces textes. Mes chers collègues, je vous rappelle que ces scrutins s'effectueront depuis les terminaux de vote. Je vous invite donc à vous assurer que vous disposez bien de votre carte de vote et à vérifier que celle-ci fonctionne correctement en l'insérant dans votre terminal de vote. Vous pourrez vous rapprocher des huissiers pour toute difficulté. Avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour le groupe du Rassemblement

deux sujets majeurs répondent à une même problématique : la dégradation d'un service public essentiel dans un État de droit. Je ferai miennes certaines des remarques formulées par mon collègue Jean-Yves Roux lors de la discussion générale.

Nos juridictions sont épuisées. Nous ne pourrons compter éternellement sur l'engagement, le courage et l'abnégation des magistrats et des agents qui les secondent au quotidien- je veux les remercier et leur faire part de notre reconnaissance.

la clarification du rôle de la justice au sein de la société, au renforcement de la première instance, à l'augmentation drastique des effectifs et à l'ouverture de la justice sur la société civile. La médiation en matière civile et plus largement les modes alternatifs de règlement des conflits

de l'activation à distance de la caméra et du micro des appareils électroniques dans les affaires de terrorisme et de criminalité organisée.

Nous sommes également favorables à la déjudiciarisation de la procédure de saisie des rémunérations prévue à l'article 17. C'est un sujet difficile, souvent marqué par des.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, après des décennies de disette et même de paupérisation, la justice de notre pays commence à retrouver des couleurs, avec un budget qui va passer de 8 milliards d'euros à près de 11 milliards. C'est une très bonne nouvelle pour les professionnels concernés, mais aussi pour l'ensemble de nos concitoyens.

Le projet de loi ordinaire prévoit près de 10 000 recrutements, dont 1 500 magistrats : c'est un progrès certain nous y veillerons. En effet, la France comptait encore, en 2022, un nombre de juges par habitant inférieur de moitié à la moyenne des pays du Conseil de l'Europe : il est urgent d'y remédier.

années. De surcroît, des attachés de justice allégeront la tâche des magistrats, leur permettant de dégager un temps précieux. Le manque d'investissement se fait également sentir en matière de places de prison. Un taux d'occupation de 120 % n'est pas acceptable. Non seulement nous avons besoin d'exécuter l'ensemble des peines qui sont prononcées, mais nous devons le faire dans le respect de la dignité humaine et de nos engagements.

Focalisés sur l'enfermement, n'oublions pas que nos concitoyens attendent aussi des résultats en matière de lutte contre la récidive. Le texte prévoit également d'améliorer l'efficacité de nos services grâce au déploiement de nouvelles techniques d'enquête.

Lors de nos débats en séance, nous avons ainsi renforcé les conditions pour procéder de nuit à des perquisitions, à des visites domiciliaires et à des saisies de pièces à conviction. Toujours en matière pénale, nous avons amélioré les droits du témoin assisté, notamment dans le cadre de l'expertise. Toutes ces dispositions étaient nécessaires pour permettre à nos forces de l'ordre de mieux lutter contre une criminalité en constante évolution, tout en préservant nos libertés.

Fréquemment dénoncée, elle ne cesse pourtant de croître d'année en année et nous en sommes en grande partie responsables. Le code de procédure pénale est l'un des symboles de cette inflation normative. La solution proposée par la commission et retenue par le Sénat est pertinente,

Nous nous réjouissons qu'une expérimentation issue des travaux du Sénat voie prochainement le jour. Le tribunal des activités économiques a le mérite de la lisibilité et de la cohérence. la cohérence. Il libérera du temps de magistrat, en confiant aux juges consulaires des contentieux qu'ils sont d'ores et déjà en mesure de traiter. Afin d'alléger des greffes surchargés, nous avons également voté le transfert aux commissaires de justice des procédures de saisie sur rémunération.

Le projet de loi organique renforce également la responsabilité des magistrats et étend la protection dont ils bénéficient à leur famille. Bien entendu, nous y sommes favorables.

sceaux d'ajouter : « Le seul levier dont nous disposons aujourd'hui, selon moi, pour faire cesser la surpopulation carcérale, consiste à construire de nouveaux établissements pénitentiaires. » Nous sommes en désaccord profond avec cette manière de gérer la surpopulation carcérale.

Je rappelle que la France a été condamnée tant en raison d'une surpopulation carcérale structurelle que pour l'absence de recours effectif permettant à un détenu de faire cesser des conditions de détention qu'un tribunal jugerait indignes.

la grande absente de ce texte. Le garde des sceaux a indiqué que des solutions étaient déjà mises en oeuvre au cas par cas, mais nous regrettons l'absence d'expérimentation officielle permettant une évaluation plus objective.

Voir dans la prison la seule punition possible, considérer la détention provisoire comme une option usuelle et non plus comme une exception et développer les comparutions immédiates conduit à remplir toujours plus les prisons. La société n'en est pas plus sûre ; les détenus et les condamnés ne sont ni mieux punis ni mieux réinsérés.

l'accès à la magistrature est l'un des aspects essentiels d'une politique de justice efficace et au service des citoyens. Nous saluons la diversification des voies de recrutement, grâce notamment à l'adoption d'un amendement de notre groupe qui facilite l'accès au concours professionnel pour les docteurs en droit.

La captation à distance de sons et d'images à partir d'objets connectés tels que les téléphones et les ordinateurs est une atteinte bien trop grave aux libertés. La suspicion sur la qualité du travail des magistrats syndicalisés est tout aussi inacceptable.

jeudi dernier, nous avons achevé l'examen en discussion commune des deux projets de loi sur la justice. Nous avons pu confronter nos points de vue et nos propositions dans un climat apaisé, ce dont je me réjouis.

Nous ne le répéterons jamais assez : c'est une mesure historique. Nous avons également habilité le Gouvernement à réformer le code de procédure pénale par ordonnance, après qu'il a rassuré la représentation nationale en apportant les garanties nécessaires ce travail de codification sera d'abord effectué par un comité scientifique, mais suivi étroitement par un comité parlementaire représentatif des groupes politiques de l'Assemblée nationale En outre, vous vous êtes engagé, monsieur le garde des sceaux, à ce que le nouveau code de procédure pénale n'entre pas en vigueur avant la ratification de l'ordonnance par le Parlement et je vous en remercie.

avions déposée en novembre 2021. Une contribution pour la justice économique sera mise en place dans ces nouveaux tribunaux afin d'inciter à recourir au règlement à l'amiable des conflits. Je me félicite également de l'adoption d'amendements déposés par mon groupe, qui tendent à associer toujours plus le Parlement à l'évaluation des expérimentations relatives aux tribunaux des activités économiques et à la contribution pour la justice économique. évidemment, nous avons avec la majorité sénatoriale quelques points de divergence sur le rôle que joueront les magistrats professionnels, sur le traitement du contentieux des baux commerciaux ou encore sur celui des procédures amiables et collectives des professions réglementées. Certes, la proposition de loi que nous avions présentée en 2021 incluait les professions réglementées du droit, mais les auditions et consultations menées depuis lors ont pu susciter des évolutions sur la question. Les débats en commission et en séance auront- je l'espère -permis de rassurer certains acteurs du monde agricole, qui avaient fait part de leurs craintes à plusieurs d'entre nous. Par ailleurs, sur l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur, dont je tiens à saluer la persévérance et la pugnacité, le Sénat a codifié la récente jurisprudence de la Cour de cassation, qui se reconnaît une compétence universelle en matière de double incrimination pour les crimes contre l'humanité. Notre groupe, quant à lui, se réjouit d'avoir pu faire adopter quinze amendements qui ont connu une issue favorable, notamment celui qui, en droit pénitentiaire, vise à mettre en place une procédure d'alternative aux poursuites disciplinaires. Concernant le projet de loi organique, nous sommes satisfaits que le Sénat ait approuvé notre proposition visant à préciser les attributions que les magistrats exerçant à titre temporaire dans les fonctions de substitut pourraient se voir confier. Par ailleurs, nous accueillons favorablement le remplacement du recueil des obligations déontologiques par une charte de déontologie des magistrats.

Je pense aux perquisitions de nuit, au recours aux moyens de télécommunication pour l'exercice des droits à un interprète et à un examen médical dans le cadre de la garde à vue ou encore à l'activation à distance des appareils connectés. Je le rappelle, ces techniques seront subordonnées à l'autorisation d'un juge et certaines d'entre elles ont d'ores et déjà cours. Permettez-moi également de regretter le rejet de trois amendements que mon groupe avait déposés et qui avaient objet le maintien de la procédure de comparution immédiate lorsque le prévenu n'est pas placé en détention provisoire, le remplacement de la référence aux conditions d'aptitude pour être assesseur de pôle social par une vérification que l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne comporte pas de mention incompatible avec l'exercice des fonctions et le rétablissement le rétablissement de l'assignation comme seule voie de saisine du juge de l'exécution en cas de contestation de la saisie des rémunérations. Pour conclure, il me semble que la trajectoire budgétaire favorable, les créations de postes annoncées

C'est également celui qu'a fait le Président de la République, en octobre 2021, lorsqu'il a décidé de lancer les États généraux de la justice, en déclarant qu'il fallait renouer le pacte civique entre la Nation et la justice et garantir l'efficacité du service public.

la réduction des délais de jugement, la volonté de transformation numérique, l'instauration d'une équipe autour du magistrat, la revalorisation de certaines professions, notamment celle de gardien pénitentiaire, les investissements immobiliers, la diversification des voies d'accès à la magistrature et l'extension du champ des infractions recevables à l'indemnisation des victimes.

reviendrai. Nous sommes donc favorables à la réécriture du code de procédure pénale par ordonnance. Certaines mesures restent peu abouties, dont la réforme de la justice économique avec l'instauration d'un tribunal des activités économiques ou l'accès à la profession d'avocat,

Dans le même temps, une saisine a été adressée par le garde des sceaux au Conseil supérieur de la magistrature, demandant que soient précisées les modalités d'exercice du droit de grève et de la liberté d'expression des magistrats, y compris sur les réseaux sociaux

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous devons prendre position sur deux projets de loi primordiaux pour la justice française. La semaine dernière, en séance, les débats ont été riches et parfois clivants ; ils nous conduisent à porter aujourd'hui un regard nuancé sur ces deux projets de loi. Commençons par les aspects que nous considérons comme positifs. En ce qui concerne le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice, le groupe CRCE ne peut que soutenir les objectifs affichés du texte, à savoir ceux d'une justice plus rapide, plus claire, en somme d'une justice moderne. Le recrutement prévu de 1 500 magistrats et 1 500 greffiers d'ici à 2027 est une réponse apportée par le Gouvernement aux importantes lacunes d'effectifs. En ce qui concerne le projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, nous soutenons bien évidemment l'ouverture du corps judiciaire sur l'extérieur, la modernisation de l'institution judiciaire, tant dans sa structuration que dans son fonctionnement, et la protection des magistrats dans le cadre de leur exercice professionnel. Aussi, nous nous réjouissons de l'adoption de quatre de nos amendements au projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice, qu'ils visent l'allongement du délai pour contester une mise en examen et une mise sous statut de témoin assisté, l'extension de la compétence des pôles du tribunal judiciaire de Nanterre

nous en avons débattu. Un recours à de tels usages est disproportionné et nous souhaitons que la procédure pénale respecte les droits de la défense. Nous voulons rappeler que, au stade de l'enquête, le mis en cause demeure présumé innocent et il convient également de souligner que le principe de loyauté de la preuve régit l'enquête et s'impose à tout agent de police. Le groupe CRCE dénonce une disposition qui n'est nullement conforme à un tel impératif et qui envoie un signal particulièrement inquiétant à tous les justiciables.

Une fois rendues acceptables pour le terrorisme, ces pratiques de surveillance seront-elles étendues progressivement à des infractions de droit commun ? C'est un risque que nous ne voulons pas négliger et nous regrettons que, par ce type de disposition, que, par ce type de disposition, le Gouvernement cherche à mettre en place une surveillance généralisée. Bien que nous ayons porté la proposition de loi de Mme Éliane Assassi visant à mettre fin à la surpopulation carcérale par le biais d'amendements, d'amendements, nous n'avons pas été entendus. Mes chers collègues, ne faisons pas l'autruche, la sonnette d'alarme a été tirée et la surpopulation carcérale atteint un niveau record : plus de 73 000 détenus pour à peine plus de 60 000 places.

Est-il vraiment nécessaire de rappeler que le respect des droits fondamentaux de tous ne doit jamais être une option et que l'emprisonnement demeure un facteur de récidive ? Il est plus que temps d'enclencher une réflexion sérieuse sur notre système carcéral. Un mécanisme de régulation carcérale, aussi contraignant soit-il, doit s'inscrire dans une réflexion globale sur la nécessité d'engager une politique carcérale réductionniste en France. Comme le souligne la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans son dernier rapport d'activité, l'inertie doit cesser. La lutte contre la surpopulation carcérale doit devenir une politique publique dotée de moyens propres et durables. Enfin, concernant

Le groupe CRCE considère que conditionner la liberté syndicale, corollaire de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion, au principe d'impartialité revient ni plus ni moins à la neutraliser.

Les événements survenus au sein du tribunal judiciaire de Mamoudzou ne sauraient suffire à provoquer une réaction législative et encore moins un bâillonnement de nos magistrats. Nous soutenons les magistrats lorsqu'ils font valoir que l'appartenance syndicale ne saurait servir de fondement à la mise en cause de leur impartialité et nous nous opposons à ce qu'une telle atteinte soit inscrite dans la loi. Le groupe CRCE considère également que l'ajout d'une charte de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l'hémicycle, n'est pas la bienvenue. Le recueil des obligations déontologiques des magistrats est suffisant. Ne les accablons pas d'obligations superflues et vides de sens.

disons-le franchement, ces deux textes ne constituent pas le grand soir de la justice. Si on peut saluer une volonté sincère, y compris en matière budgétaire, de réparer une justice qui en a bien besoin, on peut sans doute regretter que ces textes ne soient pas plus ambitieux au regard des conclusions des États généraux de la justice. Mais chaque pas est une avancée ! En ce qui concerne la magistrature, la massification du recrutement est une impérieuse nécessité. Il est primordial que nous puissions enfin avoir un nombre de magistrats et de greffiers à la hauteur des standards européens. Il y va de la qualité de notre justice, ainsi que des conditions de travail du personnel judiciaire. En ce sens, la commission des lois a fait le choix de porter à 1 800 le nombre des nouveaux greffiers au lieu des 1 500 initialement prévus. Il s'agit là de respecter le ratio entre les magistrats

la prévention de la récidive doit rester au coeur de la politique pénale. La punition ne peut se concevoir sans l'idée qu'un jour le condamné réintégrera le corps social. Réinsérer, c'est protéger société. Le projet de loi organique prévoit également d'ouvrir et de diversifier le recrutement des magistrats. C'est une nécessité si l'on veut apporter du sang neuf à l'institution et éviter l'uniformisation des parcours et des profils. Cette logique doit se poursuivre jusque dans la formation dispensée à l'École nationale de la magistrature (ENM) qui ne doit pas craindre de se confronter au monde réel, notamment aux enjeux des entreprises ou des collectivités territoriales et des élus locaux, comme le préconisait notre collègue Françoise Gatel

n'est pas question d'empêcher un syndicat de s'exprimer sur des questions d'intérêt public, ni même de confondre la fonction individuelle du magistrat avec son expression collective. à inscrire dans le texte une exigence constitutionnelle : les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Par ailleurs, l'exigence d'impartialité est aussi une exigence conventionnelle. L'exercice de la liberté d'expression syndicale n'est limité que pour autant que ces exigences constitutionnelle et conventionnelle d'impartialité seraient mises en cause. Reprendre dans la loi un principe rappelé par le Conseil constitutionnel est une mesure

Sur la question des ordonnances prévues à l'article 2 pour clarifier ou simplifier le code de procédure pénale, le groupe Union Centriste se réjouit du compromis trouvé par la commission. ne s'agit pas d'un dessaisissement du Parlement, qui conserve la mission de simplifier le code une fois que le Gouvernement aura terminé la clarification à droit constant. Cela nous paraît la meilleure solution pour fournir aux acteurs de la chaîne pénale le code de procédure pénale lisible et efficace qu'ils appellent de leurs voeux depuis longtemps. Sur l'article 3, je pense que nous sommes arrivés à une position d'équilibre, en particulier grâce à l'amendement de Bruno Retailleau qui vise à limiter la géolocalisation par l'activation d'un appareil électronique à distance aux infractions punies d'au moins dix ans d'emprisonnement.

Nous avons également exclu du champ de la captation d'images et de sons, comme le préconisait le Conseil d'État, les personnes travaillant ou habitant dans les lieux protégés, comme les cabinets médicaux, les cabinets d'avocats ou les entreprises de presse. Cet élargissement protège donc les journalistes, pour peu qu'ils appartiennent à une société de presse. Enfin, l'expérimentation relative aux tribunaux des activités économiques est évidemment une mesure positive, puisqu'elle était réclamée de longue date par le Sénat. Quant à la contribution économique, j'ai pris bonne note, monsieur le garde des sceaux, de ce que vous aviez entendu nos inquiétudes et que vous nous proposeriez des solutions afin de préserver les petites entreprises et de ne pas rendre cette justice inaccessible. Bien qu'il reste encore quelques allers-retours à prévoir,

Cette disposition, bien qu'elle ait été amendée par le Sénat, pourrait ouvrir la voie à une surveillance intrusive et généralisée remettant en question le droit fondamental au respect de la vie privée. Les garanties envisagées seront-elles suffisantes ? Privilégier la sécurité au détriment de la liberté individuelle, c'est nous orienter vers une société que personne ne souhaite. Imaginez-vous un seul instant ces instruments législatifs entre les mains d'un gouvernement extrémiste ? Nous aurons alors signé de nos propres mains l'arrêt de mort de notre État de droit. Il est impératif de veiller à ce que notre système judiciaire ne permette pas de dériver vers un État policier. Je regrette que le texte ne mette pas davantage l'accent sur l'administration pénitentiaire, la mal-aimée des missions incombant à la justice- certains d'entre nous l'ont déjà dit. Il est vrai que vous avez augmenté considérablement le budget du ministère, mais, si c'est pour construire toujours plus de prisons, votre démarche est vaine. Vous le savez autant que moi, sinon mieux : la création de nouvelles places de prison ne fera pas baisser le taux de surpopulation carcérale. La logique du « tout carcéral » n'a jamais fait ses preuves.

et plus respectueuse des droits et des libertés. Il va être procédé, dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement, au scrutin public solennel sur l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, mesdames les rapporteures, mesdames, messieurs les sénateurs, au grand soir, je préfère les petits matins qui ouvrent sur le jour. Sortir la justice de l'ornière dans laquelle elle se trouve depuis trente ans : le Président de la République s'y était engagé, la Première ministre et son prédécesseur en avaient fait l'une de leurs priorités et, personnellement, c'est une ambition que j'ai portée dès mon arrivée à la Chancellerie. Cet après-midi, c'est vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qui envoyez un signal fort à toutes les juridictions et à tous les établissements pénitentiaires de ce pays- et je vous en remercie.

Je me félicite des compromis que nous avons trouvés. Même s'il reste quelques divergences, je le dis ici : elles ne sont pas insurmontables. Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux vous dire que, selon moi, les débats font honneur à la démocratie parlementaire. Au Sénat ! Et c'est dans cet esprit de compromis et de dialogue républicain que, dès demain, je défendrai ce texte à l'Assemblée nationale.

cette définition a été fréquemment reprise par le président du Sénat, Gérard Larcher : la commune, c'est la « petite République dans la grande

face à une recentralisation, qui n'est pas seulement rampante, puisqu'elle est, en réalité, de plus en plus assumée par l'État central Les acquis fondamentaux de la décentralisation de Gaston Defferre sont aujourd'hui fortement rognés. Qu'il s'agisse des normes qui se sont multipliées,

qui ne cesse de préoccuper les citoyens qui ont accepté ce magnifique engagement au service des autres qu'est la mission municipale. S'agissant

ne nous laisse pas augurer tous les résultats que nous en attendons. Mais prenons les étapes dans l'ordre : il s'agira d'une première étape, qui n'est pas suffisante. Il y a ensuite la question de l'argent. L'autonomie fiscale des communes n'existe pratiquement plus. Le démantèlement de la fiscalité locale, par plusieurs gouvernements successifs d'ailleurs, fait que le lien démocratique par essence qu'est le lien fiscal,

bien sûr la question des dotations globales qui, après avoir été diminuées sous le mandat de François Hollande, n'ont cessé de s'éroder ensuite dans la mesure où elles n'ont jamais

projets ! Enfin, et sans revenir sur cette erreur historique qu'a été la suppression de la réserve parlementaire, qui était si utile pour les petits projets de nos communes, je veux vous dire que, si les choses s'arrêtaient là, elles seraient déjà très graves. Or elles le sont encore plus, car les communes interviennent maintenant au sein de structures qui, dans bien des cas, les empêchent d'exercer pleinement les responsabilités pour lesquelles les maires et les conseils municipaux ont été choisis démocratiquement par nos concitoyens. Les communautés de communes XXL ne sont pas seulement des périmètres décidés par voie d'autorité par l'État

et la gestion de l'assainissement, on marche sur la tête ! Ce dessaisissement des maires a une conséquence immédiate : les citoyens ne les regardent plus comme des représentants ayant la capacité de régler leurs problèmes, mais comme des personnalités qui n'exercent plus réellement le pouvoir,

situation. S'ajoute à cela le manque de respect croissant dont un certain nombre de nos concitoyens, que je ne devrais même pas qualifier comme tels, à l'égard de leur maire par leur agressivité ou leurs menaces. Le maire devient l'exutoire de toutes les frustrations de notre société, parce que, encore aujourd'hui, il est le premier visage de l'autorité. Défendons nos maires, comme nous ne cessons de le faire depuis le rapport

de maires. Il faut aujourd'hui que nous nous ressaisissions collectivement et que nous revalorisions cette fonction municipale qui est essentielle à notre vie démocratique. Le statut de l'élu doit être adapté à une fonction municipale qui, par sa complexité croissante, fait que

tirons-en les conséquences. Mes chers collègues, j'y mets beaucoup d'enthousiasme, et je vous prie de m'en excuser, mais je crois que nous abordons là un enjeu fondamental qui n'est pas correctement pris en compte. Il est grand temps, je le répète, que la France se ressaisisse pour faire vivre la démocratie municipale. La parole est

pour la démocratie locale que pour la mise en oeuvre de l'action publique. Malgré les nombreuses difficultés traversées par les maires et leurs communes, il faut rappeler cette réalité incontournable : l'échelon communal fait l'objet d'un attachement fort de nos concitoyens et reste l'échelon de proximité par excellence. Je ne peux que reprendre à mon compte le mot de Tocqueville : « Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. » Je ne cite pas Tocqueville par coquetterie. Ses mots sont profondément vrais : il y a un lien évident entre l'institution municipale et la construction de la République, car c'est dans la commune que les Français ont appris la citoyenneté et la liberté politique, qui sont au fondement de notre pacte démocratique. C'est d'ailleurs sans doute un facteur d'explication du double malaise actuel, celui des maires et celui des citoyens. Nos collègues élus se sentent dépossédés de leur capacité à influer sur le destin de la commune et de ses administrés. Nos concitoyens perçoivent, même confusément, ce sentiment de dépossession et ne sont plus sûrs de voir l'utilité de voter et de s'investir dans la vie communale. Or, dans un contexte politique marqué par de nombreuses crises, il est important que nous puissions nous appuyer sur des communes solides. Les maires demeurent les acteurs publics les mieux identifiés au niveau local. Les Français les connaissent, leur font confiance et savent pouvoir compter sur eux. La commune demeure aussi, au sein de l'architecture institutionnelle et pour les citoyens, l'échelon de proximité. Elle incarne un service public de proximité répondant à une forte demande sociale. Elle bénéficie de la clause de compétence générale lui permettant de régler par délibération toutes les affaires relevant de son niveau, sous réserve qu'elles ne soient pas attribuées à l'État ou à un autre échelon. Cela explique que les attentes à l'égard des communes soient fortes, alors que les élus s'estiment bien souvent insuffisamment armés pour y répondre, du fait de diverses évolutions, notamment le renforcement de l'intercommunalité et l'augmentation de la technicité de certaines compétences. C'est le hiatus entre ces attentes fortes et les moyens réels des communes que nous avons à résoudre ensemble pour apaiser le malaise de nos collègues élus.

proximité, subsidiarité, efficacité, initiative, projet, autant de mots que l'époque a sans doute galvaudés, mais qui témoignent bien du fait que la commune est l'échelon du faire et du bien faire. Il faut que nous capitalisions là-dessus, parce que c'est ce que nos concitoyens attendent : proximité et efficacité. Il faut donc laisser les collectivités prendre l'initiative, faire des choix, organiser la vie et les services publics locaux pour répondre au mieux aux besoins quotidiens du pays. De son côté, l'État doit consolider le rôle de la commune et du maire. En matière institutionnelle, je citerai deux exemples concrets qui sont au coeur de l'action du Gouvernement et que je me dois de vous rappeler. Le premier a trait au développement d'un véritable pouvoir réglementaire local. Pour que le maire dispose dans certains domaines d'un véritable levier juridique, loi 3DS, a consacré le pouvoir réglementaire dont disposent les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les communes, pour l'exercice de leurs compétences. doit maintenant s'en saisir pour que ce pouvoir soit mis en oeuvre plus souvent. Le second concerne l'encouragement d'une décentralisation différenciée. Les règles d'exercice des compétences locales et les architectures institutionnelles doivent pouvoir être différentes en fonction des territoires. Nous devons adapter notre organisation au

je pense au renforcement du réseau préfectoral, à l'accompagnement financier renforcé par le fonds vert, à la création d'un guichet unique de l'ingénierie

qui aura vocation à identifier des pistes pour renforcer ce soutien. Nous devons aussi tracer ensemble les grandes lignes de l'avenir de la commune pour le consolider. Nous devons soutenir les maires et pérenniser le modèle communal,

nous y travaillons avec les associations d'élus. Cela me semble indispensable pour permettre à l'action publique locale de se développer et pour apporter des réponses durables aux besoins des Français. nous devons ensemble responsabiliser nos concitoyens. Le modèle de l'électeur consommateur qui vote et qui attend ensuite tout de l'élu sans plus rien lui apporter, ni encouragement ni soutien,

Le Gouvernement dispose pour répondre d'une durée équivalente. Il aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de répondre à la réplique pendant une minute supplémentaire. L'auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute.

de la République, dite loi NOTRe, ont rigidifié l'action locale. La France communale a été particulièrement exposée à leurs effets : dilution de la voix des communes dans de grands ensembles ne correspondant pas toujours aux réalités territoriales, uniformisation des politiques, éloignement de la réalité des territoires,

Cette possibilité nouvelle permet d'articuler durablement l'action des communes et de leurs intercommunalités, en prenant en compte la réalité des bassins de vie à un niveau infracommunautaire. Cet apport est décisif pour revenir à un exercice souple et simple des compétences dans les territoires. Or, dans les faits, communes et peinent à s'approprier ce mécanisme. Ils n'en ont pas connaissance et méconnaissent la marche à suivre pour créer un pôle de proximité ou un pôle de compétences. Enfin, les services de la préfecture tâtonnent pour conseiller les maires

Symbolisant l'écoute et la proximité, ils oeuvrent dans l'intérêt général et agissent pour la République avec courage et désintéressement. La dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL) a été créée pour assurer aux petites communes rurales les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Elle est destinée à compenser plus particulièrement les dépenses obligatoires entraînées par les autorisations d'absence et les frais de formation dont bénéficient les élus locaux, ainsi que la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. La DPEL est attribuée aux communes remplissant deux conditions cumulatives : une population de moins de 1 000 habitants et un potentiel financier par habitant inférieur au potentiel financier par habitant moyen des communes de moins de 1 000 habitants, majoré de 25 %.

Ce critère apparaît parfaitement inadapté aux petites communes. Il faut le rappeler : dans notre République, la démocratie a un coût. Il paraît donc primordial que toutes les petites communes, notamment celles de 500 habitants ou moins, puissent disposer de cette DPEL. Aussi, madame la ministre, quelles mesures envisagez-vous de prendre afin qu'aucune commune de moins de 500 habitants ne soit exclue du champ des bénéficiaires de la DPEL ? Il s'agit de remédier à une véritable iniquité.

nous apparaît comme un véritable contresens historique, une rupture avec quasiment soixante ans de décentralisation, certes lente, mais qui allait toujours dans la même

Aujourd'hui, il n'est plus question de liberté. Depuis 2010, les communes doivent obligatoirement adhérer à un EPCI et, en 2015, la loi NOTRe a rationalisé la carte des EPCI par redécoupages et fusions sous le contrôle de l'État. D'un mouvement volontaire où les communes bâtissaient ensemble un projet et choisissaient les compétences concédées à leur EPCI, nous sommes passés à une contrainte et au transfert obligatoire de certaines attributions. Nombre de maires vivent difficilement ce qu'ils considèrent comme une dépossession de leurs prérogatives, d'autant plus qu'ils restent, aux yeux de leurs administrés, les premiers responsables du bon fonctionnement des services publics, qu'ils en aient ou non la compétence. Or, au regard des compétences exercées, le rôle du maire et de son conseil municipal est presque devenu secondaire derrière celui du président de l'intercommunalité. Aussi ne faudrait-il pas rééquilibrer les pouvoirs au sein des EPCI, en créant un conseil des maires dont le rôle serait de contrôler l'action de l'exécutif communautaire ?

par deux ! D'autres décisions que vous avez prises ont ébranlé un peu plus les équilibres précaires que les communes parvenaient à trouver de justesse. Je pense notamment à la suppression de la

auraient le mérite de soulager les communes. Ma question est donc simple : comment lutter contre cette évolution mortifère qui consiste à passer d'une décentralisation providence à une décentralisation pénitence ? La parole est à Mme la ministre

dite Engagement et proximité, ou encore loi 3DS, pour ne citer que ces trois exemples. À cela s'ajoute une réduction des moyens financiers qui influe sur la gestion communale, les services rendus aux populations et l'autonomie des collectivités réduction des dotations, réforme de la DGF, suppression de la taxe d'habitation et de la CVAE ... Finalement, en un peu plus de dix ans, des milliards ont été ponctionnés sur les budgets communaux. La hausse des prix et la crise de l'énergie aggravent tout cela, certaines communes n'étant même plus capables de voter un budget à l'équilibre. Presque chaque année également, de nouvelles normes sont imposées, sans concertation ni discussion préalable avec celles et ceux qui sont chargés de les appliquer : je parle ici des maires. Pourtant, grâce aux maires et aux élus locaux qui sont au plus près des populations, le couple commune-services publics est le coeur battant de la République. Faut-il rappeler comment les maires et leur administration étaient en première ligne durant le covid afin de protéger leur population ? Faut-il rappeler que, dans bien des territoires, la mairie est le seul service public qui reste, la seule porte encore ouverte pour accueillir, aider et conseiller nos concitoyens ? Tantôt des héros, tantôt mis devant le fait accompli de décisions venues d'en haut, les maires et les élus locaux ont parfois le sentiment d'être, eux aussi, les variables d'ajustement des choix et des orientations du Gouvernement. Ce manque de considération aggrave le mal-être des maires et ne permet pas à nos territoires de se développer. Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour conforter l'action des maires et garantir l'autonomie et les libertés communales ? La parole est à Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Gréaume,

est à Mme Guylène Pantel. Madame la ministre, loin de moi l'idée d'opposer les villes et les campagnes, mais force est de constater qu'un urbain vaut environ deux fois plus qu'un rural pour ce qui est du versement de la dotation forfaitaire des communes. cet écart résulte du coefficient logarithmique introduit dans le calcul de la DGF en 2005. La population prise en compte, dite « population DGF », est pondérée par un coefficient qui croît selon une progression logarithmique, de sorte que, en schématisant, un résident d'une commune de 200 000 habitants pèse environ deux fois plus que celui d'une commune de 500 habitants. On me dira que les communes rurales reçoivent d'autres aides, mais les grandes villes disposent de bien d'autres leviers encore. La raison de cet écart, on la trouve dans un rapport remis par le Gouvernement au Parlement en application de l'article 257 de la loi de finances pour 2019 : il s'agit de compenser les charges de centralité des communes les plus peuplées. Certes, on peut imaginer que le coût et l'importance des services publics sont en général plus élevés en milieu urbain, bien que la progression de l'intercommunalité ait libéré les grandes communes d'une partie de leurs charges de centralité., de centralité., la sous-densité a également un coût très important, du fait par exemple de l'entretien des réseaux de voirie ou du maintien d'équipements communaux essentiels. Dans le même temps, les petites communes doivent mobiliser des moyens pour la survie des services publics de proximité, répondre aux nouveaux enjeux de mobilité, préserver les petits commerces et, de plus en plus, prévenir des risques naturels. Lors de l'examen de la loi de finances pour 2021, le Sénat avait essayé de modifier ce coefficient logarithmique. Hélas, l'Assemblée nationale n'a pas conservé cette proposition qui, sans être parfaite, était perfectible.

Aujourd'hui, si nous voulons préserver l'avenir de nos communes, il convient aussi de conforter la relation entre le maire et son secrétariat. En effet, suivant un constat à présent bien connu dans cette assemblée, le métier de secrétaire de mairie fait partie des professions les plus en tension. Les chiffres sont sans appel : deux mille, voilà le nombre de postes à pourvoir actuellement. De nombreux départs à la retraite sont également à prévoir, un quart des agents ayant plus de 58 ans. Les causes de cette crise des vocations sont nombreuses : charge de travail, isolement professionnel, poids des normes, dématérialisation croissante, faible rémunération et absence de reconnaissance d'un statut particulier. Pourtant, le secrétariat de mairie constitue un maillon essentiel de l'ingénierie communale, puisque la plupart des démarches administratives transitent par lui, que ce soit l'état civil, l'instruction des autorisations d'urbanisme, la gestion des équipements municipaux et des opérations funéraires, les ressources humaines, la gestion du budget communal, ou encore les demandes de nombreuses subventions dont la complexité est bien connue : DETR, DSIL, fonds vert, fonds Chaleur, appels à projets, Le secrétariat de mairie est le bras armé de la politique municipale, il assure la continuité de la relation du maire avec la population de sa commune. Afin de renforcer nos communes face aux multiples défis qui les attendent, il est aujourd'hui nécessaire de rendre à ce métier sa pleine attractivité. C'est le sens des propositions qui sont faites par le Sénat, par la voix de plusieurs de mes collègues dont je souhaite saluer ici le travail. Nous examinerons d'ailleurs ce mercredi la proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, des trois rapporteurs de la mission d'information constituée sur le sujet. Améliorer l'accompagnement des secrétaires de mairie, leurs perspectives de carrière, leur formation et la reconnaissance de leur travail, voilà ce qu'attendent nos maires, en particulier dans les communes rurales, qui ont besoin d'un vrai soutien administratif et d'ingénierie. Il faut conclure, mon cher collègue ! Aussi, madame la ministre, quelles dispositions complémentaires des propositions sénatoriales le Gouvernement compte-t-il

agissons pour que les fonctions de secrétaire de mairie soient exercées à un niveau d'emploi correspondant davantage aux responsabilités exercées, à savoir celui de la catégorie B, alors qu'aujourd'hui ces fonctions peuvent être exercées par des personnes appartenant à divers cadres d'emplois, dont la catégorie C. Je veux vous dire que la revalorisation

de loi, soutenue par le Gouvernement, prévoit d'ouvrir de nouvelles voies de promotion interne, vers la catégorie B, pour les fonctionnaires de catégorie C exerçant d'ores et déjà les fonctions de secrétaire de mairie. Un autre sujet sur lequel nous travaillons d'ores et déjà nous semble également important : celui de l'opérationnalité.

des générations qui se sont succédé depuis lors a eu l'envie et l'ambition de faire, et bien faire, pour les habitants et le territoire. Or aujourd'hui, pour la première fois, nous faisons face à tant de défis pour la commune et ses élus défis posés par la complexification croissante de la mission de maire, comme ceux qui exercent leurs fonctions depuis plusieurs mandats m'en offrent un témoignage quotidien ; défis posés par un sentiment croissant d'impuissance des élus- la commune est la seule collectivité à avoir la compétence générale, mais le sentiment de limitation dans l'action est réel, à cause notamment du fonctionnement et et de la taille des intercommunalités - ; défi, enfin, de la crise civique, qui provoque une remise en cause de l'autorité, y compris au niveau communal. Tout cela peut engendrer une crise des vocations, notamment aux prochaines élections municipales,

des moyens, en fonctionnement comme en investissement, de l'ingénierie, de la simplification et de la reconnaissance : le Gouvernement et moi-même nous y employons. La parole est à M. Jean-François Longeot. M. Jean-François Longeot. Madame la ministre, je souhaiterais vous interroger sur votre vision de l'avenir des communes dans notre pays. Celles-ci constituent le socle de notre organisation territoriale et jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Elles sont profondément ancrées dans l'imaginaire français, avec l'idée bien établie de « l'église au milieu du village ». On assiste pourtant, depuis les années 2000, à une tentative de ringardisation de la commune.

Pour avoir eu l'honneur d'être maire durant près de vingt ans, je crois pouvoir dire que la commune reste indéniablement un point de repère essentiel pour nos compatriotes. Au-delà de l'attachement souvent fusionnel que l'on éprouve pour commune, cette dernière est également, notamment en milieu rural, le point d'entrée de toutes les doléances et incompréhensions de nos concitoyens. La structure communale est de loin la plus agile, comme nous avons pu le constater durant l'épidémie Malgré cette reconnaissance du rôle essentiel de la commune, il nous faut cependant être lucides : celle-ci fait aujourd'hui face à des défis majeurs. Tout d'abord, la décentralisation et la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales restent des enjeux importants. Comment peut-on affirmer vouloir renforcer la décentralisation tout en supprimant les principaux leviers d'autonomie fiscale des collectivités ? La souveraineté fiscale de celles-ci n'a cessé d'être attaquée ces dernières années.

profondément convaincue que la seule source d'efficacité des politiques publiques se trouve justement dans cette proximité si précieuse. En première ligne au quotidien, les maires permettent à nos communes de vivre et de se développer. Les témoignages de ces élus locaux quant à l'évolution de l'exercice de leur mandat doivent être entendus complexification des procédures, multiplication des interlocuteurs, lenteurs des réponses administratives, ou encore impossibilité d'anticiper le montant des aides publiques, sans oublier la perte d'autonomie fiscale ou l'oubli du principe de libre administration des collectivités locales, qui est malheureusement devenu une coquille vide. Cette complexification et cette recentralisation asphyxient l'exercice du mandat local. Pire, elles démotivent ! Désormais, un sentiment prédomine souvent, celui de la solitude et de l'impuissance des maires et des élus locaux ! Madame la ministre, comment se fait-il que, dans notre pays, la volonté de simplification se transforme en complexification, et que la multiplication des agences d'État censée aider les communes se transforme en un patchwork totalement incompréhensible ? Comment se fait-il que, là où la dématérialisation pourrait conduire à gagner du temps, elle se transforme en un éloignement progressif de l'humain, qui doit pourtant rester au coeur de toute action ? Les exemples sont nombreux : la réorganisation des finances publiques, avec un éloignement des services, mais également l'accès aux différentes dotations de l'État, avec des appels à projets qui foisonnent et une complexification, flagrante notamment dans le fonds vert Madame la ministre, quand allez-vous entendre la voix des maires qui réclament davantage de simplification et de lisibilité ? Comptez-vous regrouper les différentes dotations- DETR, DSIL,

En ce sens, le statut de l'élu est une exigence démocratique : tout citoyen doit pouvoir être candidat à une élection politique, quelles que soient ses origines sociales et son activité professionnelle. Les assemblées élues ne peuvent être le miroir parfait de la société ; néanmoins, il convient de corriger les déséquilibres les plus flagrants. Dans cet esprit, dès 1976, le rapport Guichard indiquait que la démocratie aurait peu à gagner en ne rémunérant pas, ou en rémunérant mal, les fonctions électives. Par la suite, dans la lignée du rapport Debarge de 1982, la mise en place d'un vrai statut de l'élu, qui deviendrait salarié de la collectivité,

Madame la ministre, ma question est donc très simple : le Gouvernement est-il prêt à examiner les modalités de mise en place d'un véritable statut unifié de l'élu, condition de la démocratisation des fonctions électives en France ?

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc. Madame la ministre, s'agissant de l'évolution des finances locales, le rapport public annuel publié par la Cour des comptes en 2023 est sans appel. Celui-ci souligne notamment que les dépenses des communes n'ont cessé de croître, en dépit de la place prépondérante prise par les EPCI. Ainsi, 54 % du total des dépenses de fonctionnement relevait du bloc communal en 2021. Dans le même sens, le bloc communal assume 61 % du total des dépenses d'investissement.

également l'objectif de « zéro artificialisation nette », puisque les ressources communales ne sont pas adaptées à la réalisation d'un tel objectif. Comme l'a souligné le Conseil des prélèvements obligatoires dans un rapport remis à notre commission des finances, la mise en oeuvre du ZAN va avoir un effet direct sur les rentes et la fiscalité foncières et nécessite par conséquent un changement de paradigme pour la fiscalité locale. près de deux ans après la loi Climat et résilience, le Gouvernement n'a toujours pas proposé de modèle de financement pour les contraintes liées au ZAN qui sont imposées aux collectivités locales. La France communale, c'est la France des communes qui auront très prochainement droit- du moins nous l'espérons tous -à un hectare hors ZAN ; c'est aussi la France des communes

Ces petites communes, innombrables poussières de France, rejetées dans le sillon de la comète métropolitaine, reléguées dans le « désert français », recèlent une part de notre essence nationale. Or depuis plusieurs décennies, notre pays voudrait les considérer comme un legs archaïque, un surplus de crème à gommer de notre fameux millefeuille administratif, un luxe, désormais trop coûteux. Argument fallacieux ! De l'aveu de vos services, huit petites communes sur dix avaient, en 2021, une situation financière saine. Qu'à cela ne tienne,

Or toutes les communes ne sont pas faites pour se fondre les unes dans les autres, du fait de l'éloignement géographique, des disparités sociales et économiques, de la fierté identitaire. Du reste, en dépit des incitations financières, rares furent les fusions. qui est souvent avancée reste le renforcement des intercommunalités. Or un pays ne s'administre bien que de près, et la commune, même dépeuplée ou enclavée, demeure l'échelon incontournable et le chemin le plus court vers la démocratie. Elle en est la fibre élémentaire, l'alvéole où la République prend son souffle. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si la participation électorale est toujours plus forte dans les petites communes. Leurs courageux élus sont bien souvent contraints de faire contre mauvaise fortune bon coeur. Naviguant entre des normes toujours plus touffues et chronophages et s'accommodant de moyens réduits, ils s'efforcent de maintenir un lien humain à l'heure de la désincarnation. un véritable sacerdoce municipal, presque bénévole, souvent ingrat. Madame la ministre, que veut le Gouvernement ? Veut-il une France à 10 000 communes ? Veut-il laisser dépérir ses plus petits villages pour qu'ils fusionnent, de guerre lasse ?

volontariat et lorsque cela est possible, le mouvement de rapprochement entre les communes, pour constituer des communes nouvelles. Personne ne m'a donné de consignes quand je suis arrivée ; j'ai simplement rencontré Mme Françoise Gatel ...

Nous assistons à un regain d'intérêt de nos concitoyens pour ces territoires. Certains font le choix de s'y installer pour profiter d'une meilleure qualité de vie. La petite commune n'est pas un modèle dépassé. Elle a encore de l'avenir dans notre République,

Enfin, le Sénat le rappelle souvent : il faut redonner de l'autonomie financière aux communes. À la suite de la suppression du levier fiscal, que vous avez décidée, peu de collectivités arrivent à dégager suffisamment de budget pour investir. Cette forme de tutelle déguisée est très dure à vivre pour les élus locaux, qui perdent leurs pouvoirs au bénéfice d'un grand mouvement de recentralisation qui ne dit pas son nom.

de faire naître un projet et de le financer. Ces mêmes élus nous disent qu'ils ne se représenteront tout simplement plus en 2026 ! Voilà l'état de la démocratie locale dans notre pays ! Vouloir nier cette réalité, c'est courir le plus grand des dangers. Face à cela,

Les maires attendent un peu plus de simplicité. Je vous le dis et nous vous en conjurons. Je crois que l'heure est venue de se pencher sur ce problème. Comment expliquer à un maire les

Donner des gages de confiance, c'est avancer collectivement et non pas les uns d'un côté, les autres en face ! Eh oui ! Je crois qu'aujourd'hui le temps est venu de repenser ce travail de fond, de se pencher sur les propositions que nous avons faites depuis plus de dix ans- depuis qu'un certain ministre nous avait invités à travailler sur les irritants de la loi NOTRe.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'exprime devant vous en cette fin d'après-midi tant le sujet de cette proposition de loi me tient à coeur. La restitution des restes humains a toujours figuré parmi les grands combats de mon mandat de sénatrice depuis l'affaire des têtes maories conservées au muséum de Rouen, laquelle m'avait conduite à déposer en 2008 une proposition de loi pour en permettre la restitution. Il s'est toujours agi à mes yeux d'une question de dignité de la personne humaine, de justice, de respect des cultures et de mémoire. Très bien ! Reconnaissons que les collections de restes humains ne sont pas tout à fait des collections comme les autres. Qualifiées de sensibles, elles nécessitent un soin et une vigilance redoublés par rapport aux autres pièces conservées dans les collections publiques. Comme le dispose le code civil, « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort Un certain nombre de restes humains n'ont pas leur place dans nos collections tant les conditions de leur collecte entrent en contradiction avec les valeurs qui sont désormais les nôtres. Pensons aux trophées de guerre ou à certains commerces barbares, comme celui des têtes maories. Pour satisfaire la forte demande européenne au XVIII siècle, les têtes des esclaves étaient tatouées avant d'être tranchées. Pensons aussi aux restes humains prélevés en toute illégalité à l'étranger à des fins de recherche et de documentation scientifiques. Les récits d'expéditions qui nous sont parvenus fourmillent tristement d'exemples de ces exhumations clandestines. Ce n'est pas parce que ces actions sont irréparables qu'il convient de les passer sous silence ou d'agir comme si nos collections étaient irréprochables. Il faut considérer ces restes humains comme des témoins silencieux. Engager un dialogue autour d'eux avec leur État d'origine est un travail indispensable pour rendre possible une meilleure compréhension mutuelle et bâtir des relations plus solides et apaisées. J'ajoute que, bien souvent, la présence de ces restes humains dans les collections est incompatible avec les croyances funéraires du peuple dont ils sont issus. J'en profite pour saluer Mme Gillian Bird, ambassadrice d'Australie en France, présente en tribune, dont le pays demande le retour des restes humains d'origine aborigène que nous conservons. Comme tous les Comme tous les biens appartenant aux collections publiques, les restes humains sont inaliénables. Ils ne peuvent pas être restitués sans avoir été préalablement sortis des collections, ce qui implique l'autorisation du législateur. D'où le nombre très faible de demandes de restitution auxquelles la France a accédé jusqu'ici : cinq en tout, et encore seulement deux ont été réalisées par voie parlementaire, qui est pourtant la seule juridiquement licite. Souvenons-nous de la restitution en 2020 des crânes algériens par le biais d'une convention de dépôt C'est la raison pour laquelle la commission de la culture plaide, depuis déjà plusieurs années, pour l'adoption d'une dérogation de portée générale au principe d'inaliénabilité des collections permettant de simplifier la procédure de traitement des demandes de restitution. Nous sommes en effet convaincus que notre pays a besoin d'affirmer une position claire et de se doter d'un cadre pérenne pour répondre, en toute transparence et selon des critères objectifs, aux demandes de restitution.

Le Sénat avait déjà voté en 2020 une proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques, dont l'article 2 met en place une telle dérogation. L'opposition du Gouvernement à son article 1 a malheureusement empêché la poursuite de la navette parlementaire. La commission se réjouit donc de cette nouvelle initiative, émanant d'une partie de ses membres, qui pourrait enfin permettre de lever les obstacles juridiques qui pèsent sur les restitutions de restes humains. Je veux dire combien ce texte est une oeuvre collective, madame la ministre, ce qui n'a rien d'étonnant au regard du rôle moteur que le Sénat a toujours joué en matière de restitution de restes humains. J'aimerais rendre hommage au travail de nos anciens collègues, Nicolas About et Philippe Richert, qui se sont mobilisés dès le début des années 2000 pour nous sensibiliser à cet enjeu et faire en sorte que notre pays y apporte une réponse appropriée, notamment J'aimerais aussi remercier mes collègues Max Brisson et Pierre Ouzoulias, coauteurs de cette proposition de loi, avec lesquels j'ai poursuivi ces dernières années le travail de notre commission en matière de restitution de biens culturels. Je voudrais également saluer les travaux du groupe de travail sur la problématique des restes humains dans les collections publiques,

La commission a jugé le texte équilibré pour répondre de manière satisfaisante aux différents enjeux. Le cadre législatif mis en place fixe des critères suffisamment précis et objectifs pour justifier qu'il puisse être dérogé au principe d'inaliénabilité sans prendre le risque d'une remise en cause de ce principe. Le caractère scientifique et partenarial de l'instruction des demandes permet à la fois de se prémunir contre des restitutions qui seraient le fait du prince tout en facilitant la mise en place de coopérations scientifiques et culturelles bilatérales. La commission espère que l'examen de ce texte pourra, cette fois-ci, aller jusqu'à son terme tant il répond à un réel besoin. Nous attendons du Gouvernement qu'il octroie aux établissements publics des moyens nouveaux pour leur permettre d'approfondir le travail de recherche sur leurs collections. C'est une condition indispensable pour que les dispositions de Aujourd'hui, l'identité, l'origine et la trajectoire de la plupart des restes humains conservés dans nos collections sont inconnues, ce qui empêche évidemment des pays tiers de formuler des demandes de restitution. Pour finir, la commission est consciente que ce texte n'apporte de solution pérenne qu'aux États étrangers, laissant de côté le sujet des restitutions de restes humains d'origine française. La commission est convaincue qu'il existe pourtant une problématique ultramarine nécessitant un traitement particulier compte tenu des liens étroits

C'est la raison pour laquelle la commission a chargé le Gouvernement de remettre au Parlement, d'ici à un an, un rapport identifiant des voies de restitution pérennes susceptibles d'être mises en place

Mme la ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame l'ambassadrice- merci d'être avec nous -, la semaine passée, cette proposition de loi a été examinée en commission.

Jusqu'à présent, seules deux lois d'exception ont permis d'aller au bout d'une démarche de restitution, concernant l'Afrique du Sud, en 2002, et la Nouvelle-Zélande, en 2010. Madame Morin-Desailly, c'est grâce à votre engagement et à votre combativité que ces restitutions ont pu avoir lieu. Le Sénat, sous votre impulsion, a été- on peut l'affirmer -en avance sur son temps et a ouvert la voie. Ces deux lois d'espèce ont permis des débats riches dans nos assemblées et ont contribué à faire mieux connaître ce sujet dans l'opinion publique. Grâce à vous tous, le débat est désormais arrivé Il est désormais temps de ne pas s'en tenir à des lois d'espèce, qui ne visent que des cas singuliers et qui nécessitent de revenir devant le Parlement à chaque fois, et de faire en sorte que notre droit offre un cadre clair aux restitutions de restes humains patrimonialisés, fondé- bien sûr -sur les expertises historiques et scientifiques, et sur la qualité du dialogue bilatéral. Je vous l'indiquais la semaine dernière lors de son examen en commission : cette proposition de loi n'est pas technique, elle a véritablement une dimension éthique et philosophique. Elle renvoie à notre rapport à la mort, au deuil, aux rites funéraires, à l'Histoire, à la connaissance des autres cultures

« Restes humains » : cette formule sonne étrangement à nos oreilles. On aurait pu dire « vestiges osseux », mais, dans « restes humains », il y a le mot « humain ». Quant aux « restes », ils évoquent l'importance des traces laissées et transmises. Ces restes humains ont pu entrer dans nos collections publiques dans des conditions suspectes, violentes et illégitimes. Considérés comme des trophées ou des objets de curiosité, ils étaient censés éclairer de prétendues différences entre les « races ». l'objet de trafics ou de chasses à l'homme à partir du XVIII siècle pour alimenter les théories d'adeptes de craniologie et de phrénologie, les discours scientifiques fallacieux qui ont servi de justification aux théories racistes. Dans le cas de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ce commerce ignoble a été interdit en 1831, mais on sait qu'il s'est poursuivi illégalement bien au-delà de cette date. Dès mon arrivée au ministère de la culture, il y a un an, j'ai voulu engager un dialogue avec le Parlement, notamment avec le Sénat, pour travailler ensemble sur trois lois-cadres relatives aux restitutions.

fera date. La troisième loi-cadre, relative aux biens culturels africains, nécessite encore plusieurs mois de travail et de concertations à partir, notamment, des propositions formulées par Jean-Luc Martinez dans son récent rapport. Pour en revenir aux restes humains, vous l'avez dit, ils ne peuvent pour l'instant être restitués en raison du principe de l'inaliénabilité des collections publiques. Comme je l'ai précisé en commission, il est important de rappeler que cette inaliénabilité est un principe protecteur que nous ne souhaitons pas remettre en cause. en cause. En effet, ce principe nous permet de protéger les oeuvres et le patrimoine de la Nation qui se sont transmis de siècle en siècle. En revanche, force est de constater que certains restes humains sont entrés dans nos collections dans des conditions particulièrement violentes et illégitimes. Dans ce cas, il est de notre devoir d'interroger la légitimité de leur présence dans les collections publiques. C'est tout l'enjeu du travail de recherche de provenance, qui se doit d'être rigoureux, méthodique et scientifique, et dont nous soutenons le développement. Il doit être mené par les professionnels de nos musées, qui seront de mieux en mieux formés à ces enjeux, en lien avec nos partenaires étrangers. À partir de ces recherches, grâce à votre proposition de loi, un processus de restitution pourra être engagé dans le dialogue et la sérénité. J'aimerais partager de nouveau avec vous les deux exemples que j'avais eu l'occasion de présenter en commission, la semaine dernière. Le premier exemple est celui du squelette du fils d'un chef amérindien de la communauté Liempichun, qui a fait l'objet d'une demande de restitution soutenue par l'Argentine, avec laquelle nous échangeons depuis plusieurs années. Sa sépulture semble avoir été pillée par l'équipage du comte Henry de La Vaulx, qui, entre 1896 et 1897, a parcouru la Patagonie avec l'intention, notamment, de rapporter des spécimens

il reconnaît qu'il s'agit d'un sacrilège : il se définit lui-même comme un « fossoyeur ». Il affirme : « J'ai pour moi une excuse, que diable ! car je rapporterai en France un beau spécimen de la race indienne. Qu'importe après tout que ce Tehuelche dorme en Patagonie dans un trou ou au Muséum sous une vitrine. »

voilà au moins un cas dont il nous importe désormais que des experts français et argentins questionnent la légitimité de la présence dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle. Le second exemple est celui des restes humains d'aborigènes d'Australie qui sont conservés depuis plus d'un siècle dans plusieurs musées français, notamment au Muséum national d'histoire naturelle, à Paris, et au conservatoire d'anatomie de la faculté de Montpellier. En 2014, au terme d'un long et fructueux dialogue entre la France et l'Australie, il a été décidé de mandater des experts chargés de recenser d'éventuels restes humains aborigènes figurant dans les collections des musées français en vue de leur rapatriement. Le 16 mai dernier, un comité conjoint franco-australien a pu se constituer pour trouver un accord à partir des recherches d'identification et d'authentification de restes humains qui avaient été conduites depuis 2014. Voilà à quel point le temps de la recherche peut être long, mais c'est un temps très précieux. Une fois adoptée, votre proposition de loi facilitera la restitution prochaine de ces restes humains, le processus ici décrit correspondant en tout point à ce que vous préconisez.

Vous avez également analysé les dossiers en cours d'instruction avec l'Algérie, avec l'Australie, avec Madagascar ou encore avec l'Argentine. Par vos propositions, vous réaffirmez la nécessité du dialogue bilatéral, du respect des personnes et des communautés, et de la recherche scientifique. J'y souscris pleinement et je m'engage à tout faire pour faciliter les recherches de provenance et les travaux d'identification.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, certains restes humains ont intégré par le passé de manière suspecte, voire illégitime, nos collections publiques. Parfois collectés en tant que trophées de guerre ou de conquête, ils témoignent d'un temps révolu et de pratiques anciennes qu'il ne nous appartient pas de juger. Notre rôle, en revanche, est de réparer par la loi les éventuelles injustices. Nous nous sommes récemment félicités de l'adoption du projet de loi facilitant les restitutions des biens spoliés aux familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Son examen a été l'occasion d'échanges et de témoignages d'une grande émotion en ces murs. De la même manière, notre groupe se félicite de l'adoption à l'unanimité de ce texte en commission, la semaine dernière. Il s'agit d'une loi de dignité, essentielle, qui nécessitait un espace parlementaire dédié. En effet, les restes humains sont loin d'être des biens culturels comme les autres et renvoient à des événements historiques et à des situations très spécifiques. Il était important de rendre hommage aux familles et aux États concernés par certains abus en leur consacrant une loi. J'en profite pour saluer l'engagement de longue date de Catherine Morin-Desailly, accompagnée de Max Brisson et de Pierre Ouzoulias. loi permettent une grande avancée et participent à la politique mémorielle de la France. L'accueil unanime dont cette loi a bénéficié est tout à leur honneur. Il récompense un travail de longue haleine, parfois rendu difficile par des vents contraires Cela a été indiqué lors du vote, madame la ministre : il s'agit d'un texte à dimension presque philosophique. Il touche à notre rapport à la mort et à notre manière de rendre hommage aux défunts. Cette proposition de loi permettra de simplifier et d'accélérer les procédures. En effet, comme cela a été rappelé, la nécessité de recueillir l'autorisation du Parlement avant toute restitution ralentit considérablement le processus. Cela risque de décourager les initiatives, ajoutant de la difficulté à une situation déjà éminemment complexe. Par ailleurs, le principe d'inaliénabilité protège nos collections. Des garde-fous sont nécessaires pour empêcher toute restitution irréfléchie et précipitée de restes humains intégrés aux collections publiques ; ce texte fort sécurise les procédures afin d'éviter toute dérive. L'un des amendements de notre rapporteure, adopté en commission, tend à encadrer encore davantage l'instruction des demandes.

Nos collections publiques sortiront amoindries des départs de restes humains rendus aux États demandeurs. Ces demandes pourraient s'accélérer dans les années à venir ; il deviendra alors essentiel de trouver de nouvelles manières de faire vivre ces oeuvres au sein de nos musées et dans nos territoires. Il s'agira, par exemple, de conserver des espaces dédiés au sein des salles d'exposition en s'appuyant sur des photographies, sur des animations ou sur des oeuvres numériques. Des réflexions passionnantes attendent les équipes muséales. Pour conclure, le groupe Les Indépendants - République et Territoires salue le vote favorable de ce texte et s'y associe.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je commence évidemment par saluer la constance de notre rapporteure Catherine Morin-Desailly et par féliciter les coauteurs du texte, Max Brisson et Pierre Ouzoulias, pour leur travail. Ce texte est une loi de justice, de progrès et de dignité. Ses auteurs posent les bonnes questions. Les restes humains ont une place particulière dans nos collections publiques ; de ce fait, s'interroger : le corps humain est-il un bien culturel ? L'inaliénabilité de nos collections doit-elle être un obstacle au respect de la dignité due à chaque être humain, même après la mort ? La présence de ces restes humains dans nos musées est souvent la conséquence de périodes sombres de notre histoire, de la colonisation, de l'esclavage, des guerres et du mépris des corps des hommes et des femmes qui va avec. Tout le monde a en tête la terrible histoire de Saartjie Baartman, dite, d'après les quolibets de l'époque, la « Vénus hottentote ». Née dans l'actuelle Afrique du Sud à la fin du XVIII siècle, repérée par des colons anglais en raison de sa morphologie particulière, elle a été exposée dans des cabarets anglais et français, soumise à des spectacles grotesques, humiliée, violée et asservie jusqu'à la fin de ses jours et même au-delà. En effet, de 1817 à 1974, son squelette a été exposé successivement au jardin des plantes, au Trocadéro et au musée de l'Homme. L'Afrique du Sud, dès la fin de l'apartheid, a demandé solennellement le retour de sa dépouille. Ce n'est qu'en 2002 que la France a enfin accédé à sa demande et que Saartjie Baartman a pu enfin être inhumée dignement sur la terre de ses ancêtres, 200 ans après y avoir été arrachée. Cette affaire terrible a fait bouger les lignes et le regard que nous portons sur notre histoire. Désormais, nous connaissons un vaste mouvement, compréhensible, de demandes de restitutions de biens culturels liés à ce passé, un mouvement comme je l'ai dit compréhensible, mais qui comporte des risques d'inflation législative non désirée. En effet, chaque sortie de ces collections doit être prévue Nous partageons donc le besoin d'un cadre clair et transparent pour les restitutions. Ce texte constitue en la matière une étape salutaire, le respect de la dignité des personnes étant au coeur de la démarche. Ce n'est pas la première fois que le Sénat témoigne de sa prise de conscience sur le sujet. Ainsi, la proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques, déposée par nos collègues auteurs du texte que nous examinons aujourd'hui, visait déjà à mettre en place un Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens ainsi qu'une procédure pour agir en nullité de vente, de donation ou de legs de corps humains. La navette de ce précédent texte a été interrompue puisque le Gouvernement a annoncé vouloir se saisir de la question- vous le précisiez, madame la ministre

des collections publiques après décret pris en Conseil d'État et un rapport du ministère de la culture et du ministère de tutelle de l'établissement où le corps reposait. La restitution ne pourra avoir lieu qu'auprès d'un État, qui en aura fait la demande pour un corps datant de moins de 500 ans et uniquement dans un but funéraire. Il est également prévu un comité scientifique chargé de lever les doutes en cas de problème sur l'identification des corps ainsi qu'un rapport annuel au Parlement sur les restitutions. Avec ce texte, il nous est donc proposé une solution humaine, efficace, transparente et respectueuse à la fois des États demandeurs et des principes de nos collections. Nous soutenons ce texte de justice et de dignité. La parole est

Ce texte est particulièrement émouvant parce qu'il nous rappelle des heures sombres de l'Histoire, notamment la façon dont nous avons traité les restes humains et les conditions dans lesquelles ils ont été introduits sur notre territoire. Il a été souligné une

Évidemment, la caméra de Kechiche, dans son naturalisme et dans son réalisme crus, n'épargne rien de la violence de cette scène. Il est vrai que cette histoire a changé le rapport que nous avons à la restitution des restes humains.

il est transparent et il est extrêmement précis. Il est scientifique et raisonné au travers de l'idée de solliciter l'avis d'un comité scientifique, lorsqu'il y a un doute, pour pouvoir vraiment se prononcer sur la qualification des restes humains. Madame la rapporteure, je ne peux donc que vous féliciter pour ce travail que vous avez mené de façon très rigoureuse, en lien avec le ministère de la culture. C'est pourquoi notre groupe votera ce texte.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, le temps est venu de répondre à une réalité dérangeante en reconnaissant l'histoire tragique liée à nos musées et collections publiques. Ainsi, cette proposition de loi représente une avancée significative dans le traitement des demandes de restitution de restes humains en offrant un cadre clair et transparent tout en favorisant le dialogue scientifique et culturel avec les pays demandeurs. Trophées de guerre, vols, certaines pièces de nos musées ont été collectées dans des circonstances inacceptables et incompatibles avec le principe de respect dû à la dignité de chaque individu. Tel un écho du passé, ces vestiges silencieux nous rappellent l'histoire tourmentée de l'humanité. Leur présence entre nos mains nous oblige à réfléchir profondément à la signification de la dignité humaine, à la compassion et au respect que nous devons à ces individus du passé. Il est temps de rétablir l'équilibre, de réparer les blessures de l'Histoire et d'honorer la mémoire de ceux qui ont été privés de leur droit fondamental à la dignité, même après leur mort. Cette proposition de loi, fruit d'une initiative sénatoriale transpartisane, est un premier pas crucial. En visant à autoriser le déclassement des restes humains de moins de 500 ans présents dans les collections publiques, elle représente une lueur d'espoir pour les peuples et pour les nations qui cherchent à récupérer ces témoignages du passé. La mise en place d'un dispositif-cadre dans le code du patrimoine offre ainsi une vision globale et cohérente de la restitution des restes humains. Nous ne serons plus confrontés à des décisions fragmentées et, et nous pourrons gérer efficacement les futurs cas de déclassement et de restitution tout en préservant la dignité de chaque individu concerné. allons plus loin. Pour mener à bien cette mission de justice, nous devons faire preuve de rigueur et d'impartialité. C'est pourquoi la proposition de loi tend à la création d'un comité scientifique composé de représentants des deux États concernés ainsi que des institutions détenant les restes en question. Ensemble, ils évalueront de manière précise les demandes de déclassement et de restitution en tenant compte des aspects humains, éthiques et scientifiques. collaborative et pluridisciplinaire garantira que chaque décision soit éclairée et respectueuse des individus dont les restes sont en jeu. Je salue les ajouts de la commission qui renforcent la validité scientifique des demandes de restitution. En effet, un amendement a été adopté pour empêcher la sortie des pièces avant la remise du rapport du comité mixte. Néanmoins, nous estimons que des mesures complémentaires sont nécessaires. La commission demande donc au Gouvernement de fournir des ressources pour approfondir les recherches sur les collections. La documentation sur les restes humains est primordiale pour les restitutions et pour le respect de la dignité humaine. Ce texte constitue une première étape pour les restitutions, mais n'aborde pas les restes d'origine française. Un amendement prévoir un délai d'un an pour trouver une solution pérenne pour les restes ultramarins conservés dans les collections publiques. Chers collègues, en adoptant cette proposition de loi, nous comblerons une lacune juridique majeure,

nous ne devons pas nous arrêter là. Une loi-cadre sur la restitution des biens mal acquis détenus dans les collections françaises doit suivre, témoignant de notre volonté inébranlable de faire face à notre histoire avec courage, honnêteté et responsabilité. En défendant cette proposition de loi et les amendements qui l'accompagnent, nous affirmons haut et fort notre volonté de promouvoir la justice dans la gestion des biens historiques et culturels. Ainsi, je vous appelle à soutenir pleinement cette proposition de loi et à voter en sa faveur. Nous avons l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont été oubliés, d'accorder une voix à ceux qui ont été réduits au silence et d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire où la compassion et la justice prévalent. La parole La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain a introduit dans le code civil un nouvel article 16-1 ainsi rédigé : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. » Il a été complété par la loi du 19 décembre 2008 : l'article 16-1-1 que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées [ ...] doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Nous devons à notre collègue le questeur Jean-Pierre Sueur cet ajout important. Sa proposition de loi déposée en 2005 fut une contribution majeure à la législation funéraire et à la définition du statut juridique de la dépouille mortelle. En une dizaine d'années, la loi a considérablement évolué sous l'influence de réflexions éthiques qui sont devenues prépondérantes. Le corps humain est devenu un objet de droit particulier : il ne peut être possédé et doit être traité avec dignité. Les collections publiques renferment des milliers de restes humains collectés en France métropolitaine, dans les territoires de ses anciennes colonies ou dans les pays étrangers. Leur traitement ne pouvait continuer à ignorer les évolutions éthiques et législatives qui ont conduit à la modification de notre code civil. Ces vestiges humains ont été intégrés aux collections publiques à la suite de processus historiques, politiques et muséographiques extrêmement complexes. Permettez-moi de présenter deux exemples. Le crâne de René Descartes, actuellement conservé au musée de l'Homme, fut acheté lors d'une vente par le chimiste suédois Berzelius, qui le remit à Cuvier en 1821. à Cuvier en 1821. Les os ont été déposés dans une chapelle de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. On doit sans doute cette disjonction du « chef » du philosophe à l'indélicatesse du capitaine des gardes chargé de la première exhumation du corps avant 1767. Est-il justifié que le squelette de Descartes repose pour l'heure dans deux lieux différents ? J'aimerais ensuite évoquer le destin d'un autre pensionnaire du musée de l'Homme, celui de l'assassin du général Kléber en 1800, au Caire, Soleyman el-Halabi. Empalé, il mourut dans d'atroces souffrances. Son squelette fut montré pendant de nombreuses années. Cette exposition prolongeait en quelque sorte son supplice public. Reconnaissons que cette monstration avait quelque chose de monstrueux. Il m'est agréable de souligner que c'est au Sénat, en la personne de notre collègue Catherine Morin-Desailly, que s'imposa l'idée que nous ne pouvions plus traiter les restes humains du passé avec l'indignité que nous refusons désormais aux morts du présent. Son action en faveur de la restitution des têtes maories a été exemplaire et décisive. Une méthode a été alors mise en oeuvre et elle inspire aujourd'hui la présente proposition les trois principes sur lesquels elle repose : la demande doit être instruite d'État à État ; elle doit être fondée sur un travail scientifique transparent et collégial ; et les vestiges restitués sont destinés à recevoir un traitement funéraire. Ces principes avaient été énoncés, en 2010, par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé dans un avis consacré aux problèmes éthiques posés par l'utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d'exposition muséale. Il est regrettable que les institutions muséales aient tant tardé à s'en inspirer. Gérer les collections publiques ne peut se faire sans réflexion éthique. En 2005, MM. Collinet et Metzger ont rendu au ministre de la culture et de la communication de l'époque, Renaud Donnedieu de Vabres, un rapport dans lequel ils préconisaient la création d'un comité d'éthique consultatif et indépendant rattaché directement au ministre. Après la suppression de la Commission scientifique nationale des collections, une instance de ce type pourrait sans doute assurer une réflexion pérenne sur la gestion des restes humains par les services patrimoniaux. Dans le même rapport, il était recommandé de mettre en oeuvre un plan ambitieux de récolement des collections. Près de vingt ans plus tard, il manque toujours un inventaire précis de tous les restes humains conservés dans les collections publiques. La Commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art a compétence pour s'assurer de la mise en oeuvre de l'obligation du récolement décennal prévu par l'article L. 451-2 du code du patrimoine. En élargissant quelque peu ses missions, il serait peut-être judicieux de lui confier une mission de contrôle et de coordination de l'inventaire des restes humains conservés dans les collections publiques.

Je ne sais, mes chers collègues, si vous avez fait l'expérience d'expliquer que vous alliez légiférer sur la restitution de restes humains ... Auprès d'un auditoire profane, le succès, je peux vous l'assurer, est garanti.

C'est aussi un sujet à résonance géopolitique, puisque certains de ces restes humains sont d'origine étrangère et sont réclamés par des pays tiers ou des peuples. C'est le cas par exemple, en ce moment, pour l'Australie concernant des restes humains aborigènes. Cette réalité géopolitique vient à son tour soulever un problème et un enjeu juridique. les restes humains conservés dans les collections publiques sont protégés par le principe d'inaliénabilité du domaine public. C'est exactement la même problématique que celle de la restitution des biens juifs spoliés sous le nazisme, sujet sur lequel nous avons légiféré voilà peu Toutefois, la situation des restes humains semble encore plus délicate juridiquement, dans la mesure où la procédure de déclassement n'est pas appropriée pour les faire sortir du domaine public aux fins de restitution. Car l'article R. 115-1 du code du patrimoine interdit le déclassement du domaine public des biens qui n'ont pas perdu leur intérêt public. Ainsi, nous nous retrouvons toujours face à la nécessité de recourir à la loi pour effectuer de telles restitutions, ce qui,, soulève une question de nature mémorielle et philosophique. Car déterminer les conditions de restitution de restes humains appartenant à des collections publiques interroge notre rapport à la mort, à la mémoire, et même à l'humanité. Le groupe Union Centriste, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, a été moteur pour bousculer les lignes sur cette question et faire avancer notre pays.

Il fallait donc établir une procédure générale permettant de restituer les restes humains sans mobiliser à chaque fois le Parlement. C'est bien ce que clame notre commission de la culture depuis des années. Avec le présent texte, elle sera enfin entendue. Je ne peux que saluer sa détermination, d'autant que la proposition de loi que nous allons voter a bénéficié de l'ensemble des réflexions et travaux menés sur le sujet depuis plus de dix ans. Je pense aux travaux de la Commission scientifique nationale des collections menés à la suite de la loi de restitution des têtes maories, maories, relayée par un groupe de travail pluridisciplinaire mis en place par le ministère de la culture et le ministère de l'enseignement supérieur. Ces derniers ont permis de définir les critères de restitution que nous nous apprêtons à faire entrer dans la loi qui devront être constatés par un décret en Conseil d'État du Premier ministre. Le champ du texte est restreint aux seuls restes humains identifiés d'origine étrangère. La restitution ne pourra être accordée qu'à des fins funéraires. La procédure est claire et les critères sont précis. C'est ce qu'il fallait Le texte ouvre enfin sur une dernière question qu'il faudra trancher, à savoir la restitution des restes humains ultramarins. Fidèle à son implication dans ce combat, le groupe Union Centriste veillera à ce qu'un dispositif puisse voir le jour. En attendant,

Le code civil nous rappelle que les restes humains des collections publiques ne peuvent pas être traités comme des biens ordinaires. Pierre Ouzoulias vient de le rappeler, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et « les restes humains doivent être traités avec respect, dignité et décence Le code du patrimoine les considère comme des biens publics inaliénables et imprescriptibles. Les principes d'inaliénabilité et d'intérêt public compliquent ainsi la procédure de déclassement. À ce jour, seule l'intervention du législateur permet de sortir de l'impasse. Ces dispositions restrictives font obstacle aux demandes de restitution, alors même qu'un large consensus se dégage autour de la nécessité de les rendre possibles. En 2022, le Sénat a pourtant adopté l'article 2 d'une proposition de loi définissant un cadre général de sortie. Nous pouvons regretter, madame la ministre, qu'elle soit encore dans les tiroirs du Gouvernement et de l'Assemblée nationale. Le Sénat n'a pas été le seul à évoluer sur ce sujet. Dès 1986, le code de déontologie du Conseil international des musées, reconnu par l'Unesco, a qualifié ces restes humains comme faisant partie des collections sensibles. Par ce faire, il les a exclus des collections classiques. En 2007, l'ONU a adopté une résolution inscrivant un droit au rapatriement des restes humains. En 2010, lors des débats sur la restitution des têtes momifiées maories, le législateur avait mené une réflexion sur les voies possibles pour permettre les restitutions sans élaborer des lois spécifiques. En 2018, un rapport d'enquête a été remis à deux ministères. Il dressait l'inventaire de 150 000 restes humains conservés dans 249 musées de France et 23 universités. En décembre 2020, la commission de la culture appelait de ses voeux l'adoption d'une disposition législative générale pour faciliter la restitution de restes humains à des pays tiers. Ces nombreux travaux soulignent la nécessité de cette proposition de loi. À cet égard, je salue la persévérance de Catherine Morin-Desailly. En adoptant ce texte, nous fixons un cadre juridique général attendu depuis longtemps.

En s'appuyant sur les progrès de la médecine et des connaissances sur l'évolution de l'humanité, cette proposition de loi prépare les prochaines demandes de restitutions. Je pense au groupe de travail sur l'Australie, madame l'ambassadrice. En cela, elle participe à l'amélioration constante de nos relations diplomatiques. Surtout, si un bien culturel n'est pas un bien ordinaire, les restes humains ne sont pas des biens culturels ordinaires. Au moment où notre société débat de la notion de fin de vie, nous pouvons prolonger notre réflexion au-delà du trépas et considérer les restes humains avec toute la singularité et le respect qu'ils inspirent. Cette proposition de loi nous y invite

la proposition de loi que j'ai eu l'honneur de rédiger avec Catherine Morin-Desailly et Pierre Ouzoulias a été adoptée à l'unanimité par notre commission ; elle marque l'aboutissement des travaux conduits par le Sénat sur la question particulière des restes humains.

notre pays a besoin d'affirmer une position claire et de se doter d'un cadre partagé pour répondre aux demandes de restitution en toute transparence. Car le sujet est complexe et sensible. La sortie de ces biens met en jeu le principe d'inaliénabilité de nos collections et la vocation universaliste de nos musées. Pour ce qui est en jeu aujourd'hui, les enjeux sont plus simples. Les restes humains ne sont pas des biens ordinaires. Leur restitution se justifie en vertu de principes qui sont non pas d'ordre patrimonial, mais liés au respect de la dignité des personnes et à la considération des cultures et des croyances d'autres peuples. La France a d'ailleurs déjà accepté le retour de restes humains sur la terre de leurs ancêtres par la voie législative, sur l'initiative du Sénat. À cet égard, je veux de nouveau saluer le travail de Catherine Morin-Desailly. Cependant, depuis lors, d'autres voies ont, hélas, été empruntées, au mépris du rôle du Parlement. Ce fut ainsi le cas de la remise de crânes à l'Algérie en juillet 2020, en dehors de tout cadre légal. Certes, une telle restitution correspondait à une forte attente, mais on ne peut laisser prospérer des décisions fondées sur le seul « fait du prince ». Aussi avons-nous voulu, lors de notre mission d'information de 2020, et pour l'ensemble des restitutions, fixer un cadre permettant de vérifier si la sortie du domaine public est bien justifiée et d'échapper à un traitement législatif au cas par cas. suite de ces travaux, notre proposition de loi est restée lettre morte, madame la ministre, en raison du peu d'intérêt que lui a porté votre prédécesseur, qui rejetait l'idée même d'un conseil national de réflexion. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la ligne était coupée entre le travail de fond du Sénat et une approche libérée de tout éclairage scientifique, qui était alors le choix de l'exécutif. Nous tenions en effet à ce qu'une instance constituée de spécialistes intervienne, afin de porter une analyse objective, hors de toute passion, sur l'origine de l'oeuvre, son itinéraire, les conditions de son entrée dans les collections publiques. Force est de constater que nous avons été éconduits. Les temps ont changé. Fort heureusement pour le texte que nous vous proposons, un comité scientifique, accepté par le Gouvernement, sera bien chargé d'identifier les restes humains en cas de litige. Les critères de « restituabilité » que nous proposons font d'ailleurs consensus. Il s'agit d'abord d'une demande portée par un État étranger concernant des restes humains datés de moins de 500 ans, appartenant à un groupe vivant dont la culture et les traditions restent actives, et dont les conditions de collecte portent atteinte au principe de la dignité humaine ou dont la présence dans des collections est incompatible avec la culture et les traditions

Après l'adoption à l'unanimité du projet de loi-cadre facilitant la restitution de biens culturels spoliés aux familles juives durant la période nazie, nous franchissons donc aujourd'hui une nouvelle étape. Le triptyque que vous nous aviez annoncé avance au Sénat et dans le consensus. Nous vous en remercions, madame la ministre. Vous avez ainsi annoncé un troisième texte, afin d'étudier le cas des biens culturels étrangers acquis, notamment, lors de la colonisation de l'Afrique. Nous avons, lors de notre mission, fixé des pistes concrètes et exigeantes. Le Sénat est prêt à travailler avec vous sur ce sujet plus large, mais aussi plus polémique, afin de fixer un véritable juridique en matière de restitutions, dans le respect de l'ensemble des cultures. Notre ligne sera la même éclairer l'exécutif par une analyse scientifique indépendante portant sur l'oeuvre, ses origines et son parcours, afin d'éviter polémiques, réécriture historique et fait du prince. Mais, ce soir, il s'agit d'approuver un texte que nous avons élaboré au Sénat et que vous soutenez. Madame la ministre, en vous remerciant de votre écoute et en vous redisant notre disponibilité et nos convictions pour la mise sur pied du troisième volet de ce triptyque, le groupe Les Républicains votera bien sûr cette proposition de loi. Je mets aux voix,

ce texte apparaît aujourd'hui comme une évidence - le vote à l'unanimité en est le reflet -, ce serait réduire sa portée de penser que tel a toujours été le cas. En effet, il a fallu un chemin

Les autorités françaises leur ordonnent en effet, sous peine de sanctions, de cesser la diffusion de toute publicité pour des marques de services financiers à risques. Certains organisateurs ou participants, lors d'événements sportifs

haut gauche du maillot. Ces publicités ne s'adressent pas au public français, mais les chaînes françaises ne peuvent pas intervenir techniquement ou contractuellement pour en empêcher l'apparition durant la diffusion. Le présent amendement vise donc à aménager, comme dans les cas de la publicité pour l'alcool ou le tabac, les règles de publicité relatives aux services financiers. Il y a urgence, car les téléspectateurs français pourraient se voir privés, dès septembre, de matchs européens de Rennes, Lens, Paris ou Marseille, au motif que ces équipes seraient opposées, au niveau européen, à des équipes parrainées par des marques dont les publicités sont jugées illicites en France.

pas dans un autre, ce qui pose la question de la validité des droits de diffusion de la compétition régulièrement acquis dans le pays qui n'autorise pas le sponsor considéré. Nonobstant mon admiration sans bornes pour Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame,

Je comprends que certains diffuseurs sportifs souhaitent se voir exonérés de leurs responsabilités lorsqu'ils ne font que retransmettre des images en provenance d'autres États, où ces publicités sont licites. un risque que, une fois cette dérogation admise par la loi, des annonceurs malintentionnés ne profitent de la retransmission en France pour contourner une réglementation qui protège le consommateur français. Nous avons connu cette situation, voilà quelques années, avec la publicité pour l'alcool. Les alcooliers profitaient de la retransmission en France pour contourner la loi Évin et adresser leurs publicités aux consommateurs français.

un moment donné, prenne une décision claire et explique les dispositions qu'il envisage de prendre pour lever cette insécurité juridique. Sinon,

Les évolutions technologiques et la profusion de services remettent désormais en cause la visibilité des services de télévision et de radio. La présence d'un service audiovisuel ou d'une application sur l'interface d'un téléviseur, la mise en avant d'une application sur un magasin d'applications, ou encore l'intégration d'un ou encore l'intégration d'un bouton sur une télécommande relèvent généralement d'accords internationaux entre les géants de l'internet et de l'audiovisuel, d'une part, et les opérateurs des interfaces utilisateur, c'est-à-dire les distributeurs ou fabricants d'équipements

mars 2023 la liste des interfaces éligibles au dispositif et soumis à consultation publique son projet de délibération fixant les modalités pratiques de mise en avant des services d'intérêt général. Les modifications apportées par l'article 11

Ils peuvent également exister à l'échelle locale. C'est pourquoi il paraît pertinent d'élargir la définition des SIG aux télévisions régionales ou locales. Cependant, plusieurs conditions doivent être posées. d'une condition capitalistique. Ces SIG régionaux ou locaux doivent être majoritairement détenus par l'État, les collectivités territoriales ou une personne de droit public. En somme, les capitaux doivent être majoritairement publics. Je tiens à le souligner, de plus en plus de collectivités territoriales investissent dans leurs médias locaux. Cette tendance suit celle de l'audience croissante de ces médias, les téléspectateurs appréciant ces informations de proximité, ainsi que le traitement journalistique qui en est fait. Preuve en est, les médias locaux, presse régionale comprise, sont ceux ceux auxquels les Français font le plus confiance, selon une étude de 2021. Il s'agit ensuite d'une condition liée aux missions des SIG régionaux ou locaux. Ces derniers doivent remplir une mission de service public, notamment en matière d'information. Sur ce point, il convient de rappeler que les télévisions locales signent des conventions avec l'Arcom pour émettre sur le réseau hertzien, qui comprennent des obligations de production d'informations locales sur la zone de diffusion. En d'autres termes, un encadrement très précis existe. Afin de dynamiser et de soutenir encore plus l'information locale, il est donc proposé d'intégrer les SIG régionaux ou locaux à la définition globale des SIG. L'amendement

Quant à l'amendement n° 46, il aurait pour conséquence de contredire le droit européen, qui permet aux autorités nationales d'élargir la définition des SIG au-delà des seuls médias publics. Cet élargissement à l'ensemble des chaînes de la TNT est défendu par France Télévisions afin de pouvoir peser véritablement face aux fabricants de téléviseurs connectés- c'est une évidence. Il n'y a, en effet, aucune chance

L'article 11 vise à donner une définition des services d'intérêt général pour lesquels une visibilité appropriée devra être assurée sur les interfaces utilisateur comme les téléviseurs connectés. Le présent amendement, de repli, a pour objet de préciser, pour les chaînes gratuites et privées de la TNT, les critères ouvrant droit à cette qualification, et par conséquent à leur mise en avant sur les supports connectés. Il est en effet essentiel de tenir Il est en effet essentiel de tenir compte, pour les services de la TNT qui sont assujettis à des obligations de financement de la création audiovisuelle, du niveau d'engagement dans la création, plus précisément dans la création la plus ambitieuse, à savoir la création patrimoniale- fiction, animation, documentaire de création, spectacle vivant. Un lien doit être créé entre la qualité de service d'intérêt général et l'exigence éditoriale en matière de création patrimoniale. C'est pourquoi il est proposé de réserver, pour les services privés de la TNT gratuite qui sont soumis à des obligations d'investissement, la qualité de service d'intérêt général aux diffuseurs qui se sont engagés à investir l'intégralité de leurs obligations

l'avis de la commission ? Comme cela a déjà été précisé au sujet du précédent amendement, l'objectif de l'élargissement du périmètre des SIG à l'ensemble des chaînes de la TNT est de peser par rapport aux distributeurs et aux fabricants de télévisions connectés. Il n'apparaît donc pas opportun de créer des contraintes supplémentaires qui réduiraient la possibilité d'atteindre cet objectif. La commission a émis un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Avis

l'avis de la commission ? Il n'apparaît pas utile de préciser outre mesure les critères qui seront utilisés par l'Arcom pour déterminer l'ordre d'affichage des services et programmes d'intérêt général, d'autant plus que le critère de la numérotation logique est appelé à être privilégié.

L'article 11 vise à étendre les SIG au-delà des programmes de l'audiovisuel public. Pour autant, la qualification de SIG implique, à mon sens, une certaine exemplarité dès lors qu'elle confère une visibilité particulière. Il serait difficilement compréhensible qu'une société dont les programmes portent atteinte, par exemple, aux droits de la personne relatifs à la vie privée, à son image ou à son honneur, et à sa réputation, puisse bénéficier d'une telle mise en avant. C'est

l'avis de la commission ? Il n'apparaît pas souhaitable de conditionner la qualification de SIG à l'absence de mise en demeure ou de sanction par l'Arcom, d'autant plus qu'aucune précision n'est donnée quant à la gravité des faits qui pourraient entraîner cette « double peine On peut, par ailleurs, rappeler que même France Télévisions fait l'objet de mises en demeure de la part du régulateur. Par une décision du 11 avril 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, estimant que le contenu d'un reportage traduisait un défaut de mesure dans l'évocation d'une procédure judiciaire criminelle en cours, avait ainsi mis en demeure la société France Télévisions de respecter

La manière dont est rédigé votre amendement, madame de Marco, pose quand même question puisque vous ne ciblez que le service audiovisuel privé alors que le service public peut aussi faire l'objet de mises en demeure ou de sanctions. C'est par ailleurs dès la première mise en demeure ou sanction

certains engagements chiffrés de programmation. Il en est ainsi de la proportion substantielle d'oeuvres musicales françaises ou interprétées en langues régionales, de la part des ressources consacrées à l'acquisition de droits de diffusion de films d'expression originale française, des proportions de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, etc. En revanche, il n'existe aucune obligation légale sur la proportion d'investissements dans l'information. Or l'information est pour le service public quelque chose de fondamental.

l'avis de la commission ? L'avis de la commission devrait adoucir les moeurs, puisqu'il sera favorable. La proposition consistant à obliger les chaînes d'information à investir à un niveau minimal dans l'information a été faite par le président Laurent Lafon lors des travaux de la commission d'enquête sur la concentration dans les médias. Elle a été une des rares à faire l'unanimité et à retenir l'attention de l'Arcom. L'information constitue un point fort des chaînes par rapport aux plateformes. C'est vrai ! Il apparaît donc légitime de renforcer cet avantage comparatif dans les conventions négociées avec le régulateur. Quel

on imagine difficilement contraindre une chaîne musicale, par exemple, à investir dans des programmes d'information. Il faudrait donc se limiter aux seuls éditeurs qui diffusent effectivement de l'information, mais à quel degré ? D'autre part, comment mettre en oeuvre cette mesure ?

Cet article 11 a été introduit lors de l'examen du texte en commission, sur proposition de notre collègue Catherine Morin-Desailly. Il ne nous semble pas opportun de prévoir un allongement des délais d'autorisation en vue de l'arrivée des services en

par exemple, de permettre la création d'une chaîne UHD consacrée aux jeux Olympiques de 2024. Cette disposition ne prenait pas en compte la probabilité de l'arrêt des chaînes payantes de la TNT en 2025. Or il est d'intérêt public d'innover afin d'assurer l'avenir de la TNT.

L'obligation de applicable aujourd'hui à ce mode de distribution n'apporte pas de couverture supplémentaire du territoire. Les services distribués par contournement le sont grâce au fait que le distributeur

Bargeton, pour présenter l'amendement n° 74. Les fréquences audiovisuelles appartiennent au domaine public de l'État. Les éditeurs de services n'en sont pas propriétaires et ne peuvent les céder. Contrairement au secteur des télécoms, l'usage de ces fréquences de diffusion est accordé à titre gratuit. Il s'agit là d'un élément de principe important. Dès lors, il n'est pas concevable que les opérateurs qui sont titulaires de telles fréquences puissent en tirer profit en cas de vente d'une chaîne de télévision. C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité lutter contre la spéculation liée à la « revente de fréquences » en prohibant, notamment, la cession d'une chaîne de télévision dans les cinq premières années de son autorisation par l'Arcom. Je n'évoquerai pas l'affaire ayant défrayé la chronique et impliquant une personnalité assez célèbre, qui avait valu cet encadrement voulu notamment par le Sénat.

les autorisations de nombreuses chaînes arrivent à échéance en 2025 et que l'Arcom devra en délivrer de nouvelles à cette date. Bien sûr ! C'est donc non seulement tout à fait contestable sur le fond, mais aussi particulièrement peu opportun au regard de la période qui s'ouvre. C'est pourquoi je vous invite collectivement à supprimer cet article 12.

et la confiance des citoyens dans le législateur. Bien sûr, nous nous y opposons et nous souhaitons supprimer cet article 12. Quel est l'avis de la commission ? L'adoption

Une telle disposition aurait aussi pour effet d'interdire à de nouveaux investisseurs de long terme de pouvoir concourir au développement des médias français au moment où ces derniers doivent engager des investissements considérables pour relever les défis du numérique. La commission a donc émis un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Depuis les

rend nécessaire de mesurer l'audience numérique de ces médias et jugent que l'accès aux données est insuffisant. Plusieurs plateformes refusent en effet purement et simplement de communiquer leurs données d'audience et ne rendent pas publique leur méthodologie de mesure. Du fait de

l'avis de la commission ? Les audiences revendiquées par les plateformes font rarement l'objet de publications, et leurs méthodes de calcul demeurent inconnues, ce qui constitue une nouvelle asymétrie avec les éditeurs de services traditionnels, lesquels recourent à un prestataire indépendant utilisant des modes de calcul éprouvés.

Aujourd'hui, des intérêts opposés sont en présence : ceux des producteurs indépendants, qui peuvent survivre grâce à l'exploitation de leurs droits de production, et ceux des diffuseurs, qui ont investi dans la production sans détenir de droits sur leur part de production.

dans la production constitue pour ce groupe le seul palliatif à l'absence de publicité. Alors que la BBC retire près d'1 milliard de livres sterling de ses investissements dans la production, la réglementation en vigueur en France limite ces revenus à une dizaine de millions d'euros pour France Télévisions. L'avis est donc défavorable sur ces deux

La question a été débattue au Parlement, l'Arcom s'est prononcée, et plusieurs mois de consultation et de concertation avec les acteurs ont permis de rééquilibrer les règles du jeu, en particulier entre producteurs et diffuseurs. L'accès des diffuseurs aux parts de coproduction a été assoupli, un accord interprofessionnel n'est plus nécessaire pour que les éditeurs mutualisent leurs contributions à la production, et surtout, un diffuseur peut désormais acquérir des droits sur tous les supports linéaires et non linéaires, dès lors qu'il finance majoritairement une oeuvre. de cet article contraindrait le Gouvernement à rouvrir les discussions après seulement un exercice d'application de la réforme. Elle remettrait en cause les équilibres trouvés par la négociation, qui se sont traduits par des accords professionnels entre la plupart des éditeurs et des producteurs.

de coupures publicitaires contribuerait encore davantage au délaissement de la télévision en direct au profit des contenus délinéarisés,

du nombre de coupures publicitaires a pour conséquence de réduire à la portion congrue la diffusion de fictions sur les chaînes privées en clair, puisque leur coût d'acquisition ne peut faire l'objet d'une valorisation convenable. L'instauration de cette troisième coupure publicitaire aurait par ailleurs pour effet de mieux répartir le nombre des annonces publicitaires, et donc, d'améliorer le confort du téléspectateur. J'ajoute

? L'adoption de cet amendement aurait pour conséquence de fragiliser grandement le modèle économique des chaînes privées, alors même que le coût des programmes est de plus en plus difficile à rentabiliser.

perspectives particulièrement intéressantes car elle combine les avantages de la diffusion hertzienne traditionnelle et ceux de l'interactivité permise par l'internet ouvert, ouvrant ainsi une passerelle directe entre les deux univers. univers. Alors qu'aucune barrière technologique ni juridique ne s'oppose au lancement de services, et que la très grande majorité des téléviseurs sont compatibles depuis plusieurs années avec cette technologie

les dispositions de l'article 20-5 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication permettent déjà à l'Arcom d'encadrer la reprise par les distributeurs de l'ensemble des composantes du flux hertzien émis par les éditeurs.

l'avis de la commission ? Les éditeurs de services ont aujourd'hui beaucoup de mal à obtenir des distributeurs la reprise de leur signal enrichi, comme le prévoit la norme HbbTV, preuve que le droit en vigueur est insuffisant pour corriger cette asymétrie. L'avis est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Si le

Selon l'autorité, les écrans de télévision seraient parmi les premiers responsables de l'empreinte carbone du secteur numérique en France. L'Arcep évoque même une obsolescence « culturelle » ou « marketing » qui contraindrait les consommateurs, du fait d'une logique

M. Julien Bargeton. Le, ou DAB+, est une norme de diffusion qui doit permettre de pérenniser la souveraineté du réseau hertzien terrestre de radio tout en enrichissant l'offre proposée actuellement en FM

de la FM, afin de renforcer ses audiences. Les dispositions en vigueur, prévues à l'article 19 de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, imposent d'ores et déjà l'intégration de la réception en DAB+, en complément de la FM, dans les postes de radio hors entrée de gamme et dans les autoradios équipant les véhicules neufs. Toute velléité d'étendre l'obligation d'intégration de la réception DAB+ aux équipements d'entrée de gamme et aux équipements pour lesquels la fonctionnalité radio est accessoire serait non conforme avec le cadre européen.

d'interopérabilité des récepteurs de services de radios automobiles aux véhicules neufs, dès lors que ces derniers disposent d'un équipement multimédia permettant uniquement l'accès à des services et contenus par internet. Quel est l'avis

à la FM. La généralisation de cette norme sur les récepteurs vendus aurait pour effet mécanique de ramener le prix de ce type de matériel à un niveau comparable avec le prix des récepteurs FM, selon le principe bien connu des coûts décroissants. Cette disposition n'est donc en rien incompatible avec le droit européen, contrairement à ce que soutiennent ceux qui ne souhaitent pas voir le DAB+ se développer et se substituer à la FM. L'article 15 est indispensable pour assurer l'avenir de la radio face à la

toutefois que l'amendement n° 53 n'est pas totalement compatible avec le cadre européen fixé par la directive du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. C'est assez technique et

conduit avec un flegme digne d'un animateur de la BBC. Voilà six ans que nous attendions une grande loi sur l'audiovisuel, madame la ministre. Cette proposition de loi devait permettre au Gouvernement de sortir de la torpeur et de l'inaction, qui, depuis le départ de Franck Riester du ministère, caractérisent l'action gouvernementale en matière d'audiovisuel public. Quelle déception ! ! Le départ de Franck Riester n'annonçait-il pas, en fait, la paralysie de l'action gouvernementale en matière audiovisuelle ? Il n'y aura pas de réforme de l'audiovisuel.

le cadre juridique. Le conservatisme est la règle. Finalement, madame la ministre, les critiques que vous avez formulées tout au long de cette soirée et de la précédente auraient pu être adressées à votre collègue qui est aujourd'hui chargé des relations avec le Parlement. Nos débats ont également montré que le conservatisme avait un visage, celui de tous les corporatismes et de la protection de tous les espaces de pouvoir jalousement conservés que la mutualisation progressait à la vitesse de la tortue ; que les missions du service public restaient confuses et embrouillées ; que la coopération entre les médias avançait au rythme du petit train de l'interlude d'autrefois. Qu'importe, il ne faut rien Voilà ce que la gauche, devenue la gardienne du temple, a défendu pendant toute la soirée ! Merci donc à Laurent Lafon d'avoir fait tomber les masques, et de proposer un accélérateur des indispensables mutations et de la rénovation du service public de l'audiovisuel.

Je constate également que, près d'un an après la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, aucune piste ne se dégage réellement pour satisfaire la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel. Je reste sincèrement convaincue que le modèle de taxe affectée est le meilleur moyen de garantir l'indépendance budgétaire de l'audiovisuel public sur le long terme. Il est nécessaire que celui-ci puisse remplir sereinement ses missions sans se retrouver chaque année au milieu du gué, compte tenu des débats concernant son financement. La Commission européenne l'a exprimé très clairement : l'audiovisuel public ne doit pas devenir un outil de propagande politique. Autour de nous, les choses avancent. L'Australie, le Canada et, maintenant, la Californie ont pris des mesures, par exemple pour taxer les recettes publicitaires immenses des Gafam

Celle-là est toute petite- de toute façon, je ne pense pas qu'elle pourra franchir le cap de cet hémicycle. Pour terminer,

Le service public audiovisuel est essentiel pour garantir l'accès de tous les citoyens à une information pluraliste et de qualité, ainsi qu'à des programmes culturels diversifiés.

vise à rationaliser le service public. Mon groupe y voit plutôt un risque de fragilisation de celui-ci. Ni dans le texte ni dans le débat, vous n'avez convaincu mon groupe de la pertinence d'une telle holding

dont tous les Français seraient redevables. Il s'agirait pourtant de la mesure fiscale la plus à même de garantir la plus grande indépendance de l'audiovisuel public. Au lieu de cela, vous vous êtes fait les porte-voix des chaînes privées, en demandant une troisième interruption publicitaire pour les films diffusés par ces dernières, tandis que les recettes publicitaires des chaînes publiques seraient plafonnées. Sans compensation financière garantie, de telles mesures fragiliseraient grandement les moyens de l'audiovisuel public, alors même que celui-ci a pour obligation de verser, chaque année, 500 millions d'euros d'investissements dans la création. L'audiovisuel public a besoin non pas d'une

l'enjeu principal, qui porte sur les contenus audiovisuels- que produit la télévision publique ? -peut être abordé avec plus de pragmatisme, de souplesse et d'efficacité.

Quelle sera la suite réservée à ce texte ? J'entends ceux qui, de manière péremptoire, affirment qu'il n'ira pas plus loin que le Sénat. C'est prendre bien peu en considération le travail et l'expression forte de nos collègues députés, qui, eux, ont une vision claire de ce qu'il faut faire. C'est aussi prendre bien peu en considération la complexité du paysage politique actuel, qui impose des accords. La vérité, madame la ministre, est que le changement de position du Gouvernement sur la holding, son incapacité à engager la réforme de l'audiovisuel depuis 2017 et, désormais,

plonge l'audiovisuel dans une période de flou et d'incertitude. Le Sénat, au travers de ce texte, a exprimé une vision et posé un cadre. Mes chers collègues, je suis prêt à prendre le pari que, dans quelques semaines, ou peut-être quelques mois, le Gouvernement se tournera vers le Sénat, comme il l'a déjà fait sur d'autres sujets, pour trouver une solution au problème qu'il a lui-même créé. Quoi qu'il en soit, chers collègues ! Très bien ! Mes chers collègues, en accord avec les groupes politiques, les commissions et le Gouvernement, nous pourrions, concernant l'ordre du jour du jeudi 15 juin, prévoir de commencer l'espace réservé au groupe Union Centriste dès la fin de celui réservé au groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, qui pourrait se terminer avant seize heures. Y a-t-il des observations ?